et urgent que notre assemblée puisse débattre de manière ouverte et transparente avec le Gouvernement : face aux inquiétudes de nos concitoyens, l'information la plus large sur les risques et les mesures prises

à vos interrogations, que j'imagine nombreuses, face à la menace inédite que connaît notre pays. Cette menace appelle, de la part du Gouvernement, de la rigueur, beaucoup de rigueur, et de la transparence, beaucoup de transparence. Le ministère qui m'est confié et, au-delà, l'ensemble du Gouvernement se mobilisent face à cette situation exceptionnelle. Je laisserai chacun juge de la rigueur des décisions prises et des actions engagées ; mais me voici devant vous pour la transparence. transparence. Je salue devant cet hémicycle la mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé, qui sont en première ligne, qui rassurent nos concitoyens et les prennent en charge de A à Z chaque fois que la situation l'exige, quel que soit le point du territoire national concerné. Saluer le dévouement et le professionnalisme des soignants, c'est déjà rassurer les Français. Je le dis à nos concitoyens : nous avons la chance de pouvoir compter, en France, sur les meilleurs médecins et les meilleurs soignants du monde. Et si c'est par gros temps que l'on reconnaît les bons marins, je peux vous assurer que tous les professionnels de santé que j'ai rencontrés ces derniers jours m'ont impressionné par leur réactivité, leur sang-froid et leur sens du devoir. À travers vous, je salue également tous les élus. Je sais combien ils sont sollicités, dans tous les territoires, par des citoyens inquiets pour eux, inquiets pour leurs enfants, inquiets pour leurs proches. enfants, inquiets pour leurs proches. Une crise sanitaire mondiale touche notre territoire depuis quelques semaines. Notre responsabilité collective, c'est de protéger nos concitoyens, c'est de garantir le bon fonctionnement de notre système de santé. Je vous confirme que notre système de santé est prêt et que notre vigilance est à son plus haut niveau. Depuis le 7 janvier dernier, date à laquelle le virus a été séquencé, Santé publique France mène une veille quotidienne automatique et syndromique très aboutie.

beaucoup de détermination, accomplissent un travail minutieux, en liaison avec l'ensemble des professionnels de santé de notre territoire. Le caractère global du Covid-19 requiert une coordination globale et un dialogue étroit entre les États. Nous travaillons donc en interaction avec les experts de l'Union européenne, le siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le G7 santé. Pour l'instant, et c'est heureux, nous avons réussi à nous prémunir de la machine à créer de la confusion et de la panique. Mais j'appelle chacun à la responsabilité et à la vigilance, parce que la floraison de rumeurs serait dangereuse en pareilles circonstances. C'est la raison pour laquelle nous développons une information large à destination des professionnels de santé : ces derniers jouent un rôle majeur pour faire oeuvre pédagogique. Le site DGS-urgent, destiné aux professionnels de santé, compte déjà plus de 800 000 abonnés, qui reçoivent notamment les guides et les fiches techniques régulièrement actualisés.

Les tests de diagnostic biologique dits PCR ont, quant à eux, été disponibles très rapidement grâce à l'Institut Pasteur. Par ailleurs, nous tenons des points-presse quotidiens.

Si nous assurons cette information quotidienne, c'est parce que la transparence est essentielle, parce que la situation reste très évolutive, à l'étranger comme en France. À l'heure précise où je vous parle,

quatre zones territoriales sont particulièrement touchées : une zone dans l'Oise, une zone en Haute-Savoie, une zone dans le Morbihan et une zone dans le Haut-Rhin.

Mesdames, messieurs les sénateurs, tout le monde doit montrer l'exemple, et il ne sera ni inutile ni fastidieux de rappeler devant votre assemblée les gestes qui constituent une barrière efficace contre la propagation et le risque de contracter le virus du Covid-19

appeler le 15 en cas de symptômes, ne pas se rendre chez son médecin généraliste, ne pas se rendre soi-même aux urgences ; et ne porter un masque qu'en cas de maladie- nous aurons sans doute l'occasion de reparler des masques au cours Au quotidien- je pense en particulier à la vie professionnelle -, tout le monde doit se sentir concerné. L'erreur serait de regarder ces recommandations avec détachement. Ces gestes simples sont des pratiques et des réflexes qui rendent chacun acteur de sa santé et de celle des autres. aux gestes simples, mais non aux discours simplistes. À cet égard, je rappelle que les frontières géographiques n'ont pas de sens quand il est question d'une épidémie et qu'en la matière seule compte la zone de diffusion du virus. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs utilement signalé que la fermeture des frontières ne constituait en rien une mesure de santé efficace. La semaine dernière, à

Mesdames, messieurs les sénateurs, le choix du Gouvernement, c'est d'être transparent dans l'information et déterminé dans l'action. L'enjeu, c'est la santé des Français et notre cohésion sociale. Nous vivons un moment historique ; un moment où ce que l'on croyait appartenir à un passé lointain ressurgit et interroge notre capacité collective à faire face. Nous ferons face, grâce à nos professionnels de santé, grâce au sens des responsabilités de chacun, parce que les solidarités se mesurent aussi et peut-être même d'abord dans l'adversité. L'information, l'anticipation et la prévention sont les outils les plus efficaces pour lutter contre l'épidémie. Toutes les activités essentielles à la vie des Français doivent pouvoir se poursuivre. C'est le cas dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, du recyclage des déchets, ou encore des transports. je le répète : notre système de santé est prêt à affronter cette épidémie, mais la mobilisation de chacun est requise. Cette mobilisation permettra de ralentir la propagation du virus, et donc de limiter les effets de cette épidémie sur le fonctionnement de notre système de santé et sur la vie de nos concitoyens. Il y a une inquiétude en France. Cette inquiétude est légitime. Je l'entends, je la comprends et j'y apporte quotidiennement le maximum de réponses. Nous sommes prêts, nous sommes mobilisés et nous avons plus que jamais l'esprit de responsabilité qui permet de vaincre toutes les menaces ! La parole

Dans la lutte contre l'épidémie, l'information fait partie de nos armes. Informer les soignants, les patients, nos concitoyens, prévenir les rumeurs, démentir les fausses nouvelles : ce débat peut y contribuer et, mieux informés, nous pourrons être plus utiles encore. Nous connaissons encore peu de choses du coronavirus, émergeant depuis deux mois, même si le séquençage de son génome a été réalisé avec une grande rapidité, ce qui a permis de l'apparenter à des virus connus, comme le SRAS. La faiblesse de nos connaissances peut susciter beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup de craintes. Ces craintes sont légitimes. Oserai-je dire qu'elles sont nécessaires dans la réponse à l'épidémie En effet, des virus mieux connus n'en sont pas moins dangereux. Chaque année, dans notre pays, on meurt par milliers de la grippe saisonnière, ou encore de la rougeole, alors qu'une réponse vaccinale existe et que les gestes barrières peuvent protéger.

en protections contre le virus. Nous savons qu'un réservoir de virus émergents existe, et qu'il est même très important. Nous devons vivre avec ce risque l'accélération des contacts et des échanges, la fréquence des déplacements, le rythme croissant des mobilités sont des chances, mais ils favorisent aussi la propagation des virus. Quel est l'état des connaissances sur le coronavirus en 2020 ? Que savons-nous de ses caractéristiques et de la façon dont il se transmet ? Y a-t-il un danger de transmission mère-enfant ? Que savons-nous des possibilités de mutation ? Il ne semble pas que l'on ait observé de mutation jusqu'à présent, mais ce facteur serait un élément décisif dans la réponse à apporter. Les traitements aujourd'hui dispensés aux patients sont transposés d'autres pathologies, en particulier du VIH. D'autres pistes ont été avancées sur le fondement d'essais cliniques effectués en Chine. Que penser de la qualité de ces essais ? La chloroquine, déjà évoquée dans d'autres indications et pour des épidémies précédentes, est-elle une piste ? Nous nous interrogeons sur les traitements, mais aussi sur les vaccins. Un vaccin est-il à notre portée si l'épidémie se prolonge ? Dans quels délais pourrions-nous en disposer ?

Elle suppose aussi de mieux impliquer les professionnels de la médecine de ville, qui se sentent encore insuffisamment armés dans la réponse au virus et trop peu informés quant à sa prise en charge.

Même si nous connaîtrons sans doute des victimes jeunes et bien portantes, comme pour la grippe, le coronavirus est plus létal pour les personnes âgées. Ne devons-nous pas en tirer des conséquences sur le port du masque et sur l'accueil et sur l'accueil dans les Ehpad de notre pays ? Nous avons donc beaucoup de questions et j'espère que le débat permettra d'y répondre. Je souhaite aussi qu'un point régulier puisse être organisé devant la commission des affaires sociales, afin que ses membres puissent se faire les relais, au sein du Sénat et dans leurs territoires, d'une information au plus près des derniers éléments disponibles. Les précédents nous montrent que la réponse des pouvoirs publics est toujours critiquée : l'épidémie est ravageuse, on lui reproche son incurie qu'elle soit moins offensive que prévu et on lui reprochera d'en avoir trop fait ! Informer au jour le jour, admettre que l'on ignore certaines choses, développer la culture du risque favorise la résilience de la population et prépare notre pays à des crises qui se répéteront forcément. Le quotidien a fait état de l'augmentation des ventes du livre d'Albert Camus,, à la faveur de l'épidémie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'épidémie de coronavirus qui s'étend davantage sur notre territoire jour après jour aura au moins le mérite d'imposer le présent débat. Celui-ci est censé porter sur les mesures de santé publique visant à combattre l'épidémie. Il eût été préférable que le Gouvernement adopte les dispositions utiles voilà plusieurs semaines, plutôt que de tenter de dissimuler ses responsabilités derrière un débat dont nos concitoyens n'ont que faire. Les Français souhaitent des actes et non de vaines paroles. Certes, il y a eu des actes symboliques, destinés à la communication de l'exécutif, comme le confinement des enfants de retour d'Italie. Dans le même temps, pourtant, des milliers de supporters de football italiens déambulaient dans les rues de Lyon. Il y a eu aussi des mesures prises, toujours à des fins de communication, la dernière en date étant d'interdire les rassemblements de plus de 5 000 personnes. Belle réussite ! Nous avons appris ce jour que, parmi les 2 000 personnes ayant récemment participé à un congrès évangélique à Mulhouse, les services sanitaires déploraient déjà dix nouveaux dix nouveaux contaminés. Le nombre d'individus atteints croît donc de jour en jour. Peut-on vraiment s'en étonner ? Démontrant son impéritie, le Gouvernement n'impose toujours pas un contrôle thermique des personnes revenant des zones à risque. Nos aéroports voient librement circuler des voyageurs sans que quiconque s'intéresse à leur état de santé. Si l'on voulait favoriser la propagation de l'épidémie, nul ne s'y prendrait autrement. Pourquoi l'exécutif n'a-t-il pas mis en place une procédure visant à assurer la traçabilité des personnes issues de pays connaissant eux-mêmes les affres du coronavirus ? Sans cette disposition, il est impossible de suivre les individus potentiellement dangereux. C'est là une marque de l'irresponsabilité gouvernementale. Tout aussi irresponsable est la décision de ne pas rétablir un contrôle à nos frontières, mais il est vrai que la santé de nos concitoyens ne justifie pas que l'on s'affranchisse du dogme de la libre circulation, si cher à la Commission européenne ! Ce libéralisme incontrôlé a également induit la délocalisation des productions des principes actifs médicamenteux vers des pays frappés de plein fouet par cette épidémie. Aujourd'hui, nous encourons une pénurie de médicaments, car 80 % d'entre eux sont produits désormais en dehors de France et d'Europe. Je ne puis oublier d'évoquer la pénurie de masques, utiles à nos personnels de santé, dont certains se sont vu proposer des produits périmés. Pour clore toutefois sur une note moins sombre, pourrions-nous savoir si les perspectives de traitement offertes par la chloroquine contre le coronavirus sont à la hauteur des attentes de tous ? Qu'en est-il également d'un futur vaccin ? La sagesse indique que gouverner, c'est prévoir. Il est patent que le Gouvernement a sous-estimé l'ampleur de cette épidémie, en négligeant la mise en oeuvre rapide de dispositions pourtant élémentaires. Cette gestion de crise au doigt mouillé est révélatrice de la désinvolture de l'exécutif ; les Français en paient aujourd'hui le lourd tribut.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux commencer mon intervention en saluant le dévouement des personnels hospitaliers qui effectuent un travail remarquable, au moment où la France est le deuxième foyer d'infection du coronavirus en Europe, derrière l'Italie. Malgré la diminution constante des moyens depuis des années, notre système hospitalier continue à prendre en charge les malades avec un esprit de responsabilité, grâce à l'engagement des personnels soignants et administratifs. Je tenais une nouvelle fois à le souligner en mon nom comme au nom de mon groupe. monsieur le ministre, au-delà des compliments que vous leur avez adressés, quelles mesures concrètes prenez-vous en leur faveur ? Compte tenu de la vitesse de propagation du Covid-19, le passage au stade 3 de la lutte contre l'épidémie semble n'être plus qu'une question de jours. Le Premier ministre a invité jeudi 27 février, en votre présence, les responsables des partis et les présidentes et présidents des groupes parlementaires, afin de faire le point de la situation et de partager les informations dans la plus parfaite transparence. C'était une sage décision. J'y représentais le groupe CRCE, à la demande de sa présidente, Mme Éliane Assassi. Des idées, des suggestions, des propositions vous ont été faites, mais je n'ai pas l'impression qu'elles ont été suivies d'effet. Permettez-moi donc d'avancer quelques remarques. Comme l'a justement souligné M. Fabien Roussel, secrétaire national du parti communiste français et député du Nord, il n'est pas dans notre intention d'instrumentaliser cette question de santé publique à des fins politiciennes. Cette remarque vaut pour tout le monde : permettez-moi de dénoncer le choix du Premier ministre, à la faveur d'un conseil des ministres convoqué en urgence et consacré exclusivement au coronavirus, d'avoir dégainé le 49-3 à propos d'une question d'intérêt général, notre système de retraites. Revenons à vos décisions. Vous avez ouvert un numéro vert, ce qui est une bonne mesure. Pourtant, monsieur le ministre, pour que le service rendu soit optimal, il ne faut pas que le standard soit saturé en journée ou que le numéro ne soit pas joignable après dix-neuf heures, ce qui est malheureusement le cas, faute de personnel en nombre suffisant ! Vous avez également pris la décision d'annuler tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné et dans certains milieux ouverts, en cas de risques de contacts avec des personnes et de circulation possible On sent monter un climat anxiogène, d'autant que des rumeurs infondées se répandent les réseaux sociaux. La meilleure riposte est donc la transparence, la diffusion régulière d'informations, comme dans le cadre des réunions organisées par les préfets, ou encore les conférences de presse quotidiennes que vous tenez. C'est ce que fait le Gouvernement ! Cependant, monsieur le ministre, ce qui peut faire la différence, ce sont les moyens humains et financiers mis à disposition de l'hôpital public et les mesures d'accompagnement pour la médecine de ville. Or, depuis un an, les personnels soignants conduisent une action pour dénoncer la crise que vit l'hôpital, à la suite des politiques de restrictions budgétaires mises en place depuis des dizaines d'années et accentuées par Mme Agnès Buzyn. Les grèves, les mouvements unitaires allant des aides-soignants jusqu'aux chefs de service ont dénoncé, et continuent de le faire, la politique dévastatrice pour notre système de soins que mène votre gouvernement. Faut-il rappeler les chiffres et la suppression de 1 milliard d'euros pour les hôpitaux publics en 2020 ? La ministre Mme Agnès Buzyn leur a concédé 300 millions d'euros, soit un manque à gagner de 700 millions d'euros pour revenir au budget initial, mais pas pour résoudre la crise. Monsieur le ministre, comme Mme Buzyn, vous semblez aimer le jeu de bonneteau : vous annoncez « débloquer 260 millions d'euros d'aides pour les hôpitaux », mais, détail important, ce soutien financier sera pris sur les « réserves de l'exercice budgétaire 2019 non dépensées », autrement dit, sur le budget de l'hôpital

Le directeur général de la santé a tenté de nous rassurer sur la disponibilité de 2 400 lits de soins intensifs et de réanimation dans les 108 établissements dédiés. Où vont aller les patients qui occupent aujourd'hui ces lits pour d'autres pathologies ? Rappelons qu'avec les groupements hospitaliers de territoire (GHT) de nombreux hôpitaux de proximité ont été vidés de leurs missions par des fermetures de services et des suppressions de lits. Vous nous dites que vous éprouvez des difficultés à recruter des infirmières et des aides-soignantes. Répondez donc à la revendication des personnels

qu'ils l'ont dit, qu'ils l'ont crié, rien ne change ! Il faut au moins 100 000 embauches sur trois ans, une revendication que nous avons reprise dans notre proposition de loi pour faire face à l'urgence de la situation des Ehpad. Pour le moment, nous n'en constatons aucune ! Comment les personnels des Ehpad pourront-ils répondre à vos préconisations, monsieur le ministre ? « On veut bien plus de masques, mais encore faut-il avoir des personnels pour les porter », a ainsi déclaré, à juste titre, M. Patrick Bourdillon de la fédération CGT de la santé. Il faut donc des préconisations, oui, de l'information, oui, de la transparence, oui,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, combien de temps l'épidémie va-t-elle durer ? Combien fera-t-elle de victimes ? La réponse technique et précise à ces questions est la suivante : Dieu seul le sait Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos dirigeants, en ces temps où la défiance est devenue une religion nationale, aggravée par les réseaux antisociaux, amplifiée par le complotisme. La science avance trop lentement pour nourrir les télévisions de l'immédiat, qui lui imposent une épreuve redoutable. Il faut informer sur la propagation au jour le jour, expliquer les mesures mises en place alors que la situation change sans cesse, annoncer les aggravations progressives sans déclencher de panique. C'est la lutte de la raison contre l'émotion ; or, dans le monde d'aujourd'hui, la seconde part malheureusement favorite. Pour inverser la donne, nous pouvons compter sur un système de santé préparé, coordonné et supervisé avec fermeté et souplesse, et sur des professionnels de santé qui sont les rares à bénéficier encore, à juste titre, de la confiance de nos concitoyens. Nous pouvons compter aussi, à ce jour, sur l'attitude responsable des principaux partis politiques, choisissant la solidarité et la confiance dans dans les équipes soignantes plutôt que de chercher ce que le Gouvernement aurait pu faire de travers. Bien sûr, l'exception que l'on attendait s'est produite, nous venons d'en avoir ici même la démonstration. Je parle de ceux qui ont sauté sur l'occasion pour ressortir des cartons leur obsession de la fermeture des frontières. Trente ans après le ridicule de ceux qui avaient annoncé que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté sur le Rhin, on aurait pu espérer échapper à ce genre de suggestions. Rappelons donc aux partisans de la ligne Maginot virologique que les micro-organismes circulent sans visa. Au XIV siècle, à un moment où la lenteur des transports freinait mille fois plus les déplacements que la plus stricte fermeture possible des la peste venue d'Asie a tué le tiers de la population européenne après avoir franchi toutes les barrières. Les chiffres d'aujourd'hui ou de demain n'ont rien à voir avec cela. Des mesures précises, adaptées, conformes à l'avis des spécialistes, doivent être prises, même lorsque certaines d'entre elles sont pénibles. La responsabilité du Gouvernement est que la précaution l'emporte sur la psychose, le contrôle maîtrisé sur le blocage du pays et la réponse sanitaire sur les emportements idéologiques. une deuxième réflexion : depuis la chute des bourses et la baisse en catastrophe du taux directeur de la Réserve fédérale américaine, tout le monde a compris que la crise économique mondiale à venir risquait d'être aussi grave que la crise sanitaire, je n'insiste pas. Je veux toutefois rappeler une vérité inquiétante : pour des produits d'importance vitale, tels que les médicaments, nous sommes devenus dépendants d'un seul pays, la Chine. Quand ses usines ferment parce que la population est consignée, la production s'arrête. L'an dernier, mon groupe, sur l'initiative de M. Jean-Pierre Decool, a lancé un cri d'alarme en créant une mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins. Celle-ci a établi qu'il était suicidaire de ne dépendre que d'un seul fournisseur. L'époque où l'on achetait tout là où les coûts étaient les moins élevés est révolue en ce qui concerne les productions stratégiques. L'aspect positif de cette crise est peut-être de révéler clairement qu'il est temps d'agir. Les changements seront difficiles, il faut les préparer. Ma troisième réflexion est que, à l'heure où certains sont séduits par les régimes autoritaires, le jeune médecin de Wuhan, devenu un héros, nous a rappelé, avant sa mort, qu'après le virus le principal responsable de la pandémie était la dictature chinoise. Le mois et demi perdu par la peur du régime d'apparaître pris au dépourvu et par la terreur des autorités locales d'être châtiées pour un événement dont elles n'étaient pas responsables a fait perdre la première bataille, celle qui aurait pu tout stopper. C'est une tragique ironie de voir ce pays, dans lequel chaque habitant est épié en permanence par des caméras, passer pendant cinq semaines à côté d'une épidémie évidente. Les dirigeants chinois en ont-ils tiré la leçon pour aller vers plus de démocratie ? Évidemment non, au contraire : on va vers encore plus de censure et de répression. Je ne serais pas surpris d'apprendre que la prochaine mesure- je ne suis même pas sûr de plaisanter -soit d'adjoindre aux caméras optiques de chaque rue des caméras thermiques pour punir les criminels qui oseront désormais sortir de chez eux sans avoir pris leur température. Je terminerai en disant que si je parle au nom de mon groupe ce soir, c'est parce que je suis médecin épidémiologiste. J'ai commencé ma carrière en Inde au XX siècle, au moment de la campagne d'éradication mondiale de la variole, cent fois plus mortelle que le coronavirus. À l'heure actuelle, les moins de 25 ans n'ont plus sur le bras la cicatrice gaufrée qu'ont tous ceux de nos générations, parce qu'on ne vaccine plus contre la variole : le virus a disparu de la surface de la Terre. C'est un nouveau combat que le monde doit gagner aujourd'hui. Le Sénat est à vos côtés, monsieur le ministre, aux côtés de tous nos professionnels de santé et aux côtés de tous nos concitoyens dans l'épreuve que nous traversons et que, bien entendu, nous surmonterons.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Face à un climat anxiogène, je me félicite de la tenue de ce débat sous la forme de questions-réponses. Il permettra de rétablir quelques vérités quant à la situation actuelle.

Selon le centre chinois de contrôle des maladies, 80 % des cas d'infection sont considérés comme bénins. Le taux de létalité du nouveau coronavirus est relativement bas

Enfin, l'indice de contagiosité du virus est lui aussi relativement faible, entre 1,5 et 3,5. À titre de comparaison, celui de la varicelle est de 8,5 et celui de la rougeole de 9. Ce n'est pas parce qu'un virus a un indice de reproduction et une létalité faibles qu'il est inoffensif. La grippe saisonnière est dans ce cas de figure pour la saison 2018-2019, elle a fait 8 100 morts en France. Le Covid-19, de son côté, a tué à ce jour plus de 3 000 personnes dans le monde, dont quatre Les médias ont donc un grand rôle à jouer dans la gestion de cette situation sanitaire. Moins de sensationnalisme et davantage de messages de prévention sont une partie du remède. Ces messages ont été rappelés par le ministre. Le Gouvernement doit également faire preuve de clarté et d'une grande pédagogie dans l'explication de son plan de gestion du risque. Certaines incohérences, au moins certaines décisions perçues comme telles, dans la mise en oeuvre des actions d'endiguement sont pointées du doigt pourquoi annuler le semi-marathon de Paris et non certains matchs de football ? C'est une question de proportionnalité, je l'entends bien, mais nos concitoyens ne le comprennent pas toujours. Chaque Français Chaque Français est, enfin, responsable des informations qu'il véhicule. Chacun d'entre nous peut participer, à son insu, à l'installation d'un climat anxiogène contre-productif. L'une des conséquences les plus préjudiciables en serait la saturation des hôpitaux. Les professionnels de santé- je veux également les saluer -se préparent, dans un contexte particulier pour l'hôpital public. Il y a quelques semaines, plusieurs centaines de chefs de service ont démissionné de leurs fonctions d'encadrement pour dénoncer le manque de lits et d'effectifs. Différents plans gouvernementaux se sont succédé ces derniers mois, sans jamais emporter la pleine satisfaction des personnels hospitaliers. Aussi, je me félicite que le Gouvernement ait débloqué 260 millions d'euros supplémentaires issus de la mise en réserve prudentielle pour faire face à cette situation. Je regrette néanmoins que l'hôpital public bénéficie d'enveloppes supplémentaires au gré des situations de crise et non de façon pérenne et programmée. De l'aveu de médecins, certains hôpitaux sont déjà débordés, alors que le nombre de patients hospitalisés est encore faible. L'un des enjeux sera de maintenir un niveau de soins élevé pour les personnes hospitalisées pour d'autres motifs que le coronavirus. Enfin, face à un système hospitalier en difficulté, il nous faut éviter la contamination du personnel soignant.

Face à l'actualisation en continu des instructions ministérielles, ne faudrait-il pas une communication commune, unique à l'échelon national, pour l'aide à domicile avec des déclinaisons locales selon l'intensité de l'épidémie dans chaque département ?

L'OCDE a ramené sa prévision de croissance planétaire de 2,9 à 2,4 % pour 2020. Celle-ci pourrait même être divisée par deux en cas d'allongement de la durée de l'épidémie. Le risque de récession est désormais envisagé. La France est également touchée : la croissance nationale pourrait passer sous les 1 % cette année. Pour conclure, le coronavirus met au défi notre société mondialisée. Il révèle les failles de nos systèmes d'organisation. Il conduit à s'interroger sur les fondations de nos systèmes économiques.

Merci

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour débattre des mesures de santé publique prises, et à prendre, pour éviter la propagation du coronavirus en France. Innover sur ce sujet paraît bien difficile, tant les informations et les commentaires plus ou moins scientifiques inondent nos chaînes d'information depuis maintenant plusieurs semaines. Cela ne doit toutefois pas nous exempter d'un débat sur le fond, loin de certaines polémiques politiciennes qui se nourrissent de chaque crise pour prospérer, comme un virus sur sa cellule. Nous en avons eu un triste exemple dans cet En ma qualité de médecin, je m'efforce de considérer avant tout les faits, de les appréhender de manière scientifique et pragmatique. Les faits, ce sont plus de 250 malades

Néanmoins, bien que nous en soyons au début de l'épidémie, le bilan du Covid-19 est très loin de celui de la grippe, qui, chaque année, contamine 2 à 6 millions de Français et en tue plusieurs milliers. Je fais ce parallèle en espérant que la prise de conscience que nous connaissons aujourd'hui infusera dans la société pour les hivers à venir. Je n'aurai de cesse de le répéter : la prévention doit être au coeur de notre politique de santé publique.

Se vacciner, c'est se protéger, mais aussi protéger ses proches, notamment les plus fragiles, qui paient plus lourdement les conséquences de ces maladies. C'est pourquoi nous devons, ensemble, continuer de militer pour une généralisation de la vaccination, notamment parmi les professionnels de santé, dont seulement 25 % se font vacciner, alors qu'ils sont en contact direct avec les populations les plus fragiles. En matière de prévention, je salue, monsieur le ministre, les mesures prises par le Gouvernement pour réquisitionner la production française de masques et la réserver en priorité aux professionnels de santé et aux malades

à formuler. D'abord, la population a pu avoir le sentiment que l'État, peut-être, avait réagi aux événements un peu tard. N'aurait-il pas fallu mettre en place des mesures de réquisition et de délivrance sur ordonnance des masques dès les premières contaminations françaises ?

certains pharmaciens continuent d'indiquer qu'ils ne disposeront pas de quantités suffisantes pour fournir l'ensemble des professionnels de santé concernés. À ce sujet, des doutes subsistent : monsieur le ministre, pouvez-vous rassurer

S'agissant des masques, le plus gros fournisseur de France a indiqué que 70 % de sa production était basée en Chine, et qu'il ne pouvait plus rien recevoir depuis deux mois. La production française a donc été dopée et réquisitionnée : c'est fort bien, mais il est probable qu'elle ne suffise pas à pallier des décennies de dépendance croissante. l'élaboration duquel j'ai participé, a avancé plusieurs propositions invitant les pouvoirs publics à engager rapidement des mesures pour relocaliser la production de médicaments en France, ou plutôt en Europe.

à l'information sur les gestes de bon sens, qui semblent bien intégrés par la population, et à la limitation des rassemblements que vous avez décidée, on peut espérer contenir, voire limiter, la diffusion du virus. à l'efficience de notre système de santé, dont il faut saluer les grandes qualités, à commencer par l'engagement de ses professionnels, on peut aussi espérer contenir les conséquences les plus graves de la maladie.

est à M. François Patriat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, convoquer, la semaine dernière, une réunion des responsables des différents groupes politiques et des chefs de parti

Nous donner, ce soir, l'opportunité d'un débat public sur l'action du Gouvernement est primordial pour l'information de nos concitoyens, gage de transparence et de responsabilité.

Une prise en charge globale de la situation nécessite une réponse en matière de sécurité sanitaire, bien entendu, mais aussi des mesures sociales, économiques et numériques, et bien d'autres

l'Organisation mondiale de la santé a alerté du risque d'une potentielle pandémie, à la suite d'une multiplication des zones touchées par le coronavirus. À ce stade, quatre-vingts pays ont signalé des cas à l'intérieur de leurs frontières.

Reste qu'il ne faut rien sous-estimer. Si la propagation du virus à l'échelle internationale est d'une grande rapidité, nous ne devons pas non plus céder au catastrophisme. Il faut préciser que, dans près de 81 % des cas, cette maladie est largement bénigne. À l'occasion de l'irruption du Covid-19 en France, les autorités sanitaires ont enclenché le stade 2 du plan de prévention et de gestion, visant à freiner la propagation Par les actions menées, nous retarderons aussi longtemps que possible le passage au stade 3, correspondant à la circulation réelle et large du virus à l'intérieur du territoire. Mais en cas de passage à ce niveau, monsieur le ministre, quelles restrictions pourraient être mises en oeuvre ? Par ailleurs, un suivi des personnes s'étant rendues dans des zones à risque a été assuré, et des règles de réduction de la vie sociale leur ont été justement imposées. Un décret du 31 janvier dernier prévoit le versement d'indemnités pour arrêt de travail de vingt jours, sans délai de carence ; cette mesure sociale bénéficie également aux parents des enfants dont l'établissement scolaire fait l'objet d'une fermeture temporaire et qui ne peuvent se rendre au travail. Les Les évoqués par M. le ministre ont été rapidement détectés. Des mesures raisonnables, mais néanmoins contraignantes, ont été prises au moment opportun. C'est ainsi que certains événements ont été reportés à la suite de décisions locales, dans un souci de prévention de possibles nouvelles contaminations.

nous savons que la réponse sanitaire doit être territorialisée, en métropole comme en outre-mer. Afin de transmettre les recommandations adéquates et de répondre aux inquiétudes légitimes des citoyens, les préfets, les agences régionales de santé (ARS), les professionnels de santé et les élus locaux collaborent en bonne intelligence. Cette gestion se caractérise par la diffusion d'une information transparente, régulière et de qualité à destination de la population. Ce qui paraît indispensable, compte tenu du nombre de rumeurs qui se propagent sur internet. D'ailleurs, le Gouvernement a tenu avec les principaux moteurs de recherche une réunion Les Français ont confiance dans notre système de santé et dans sa gestion des crises sanitaires. À ce titre, je salue à mon tour l'ensemble les professionnels qui, aujourd'hui comme hier, se dépensent sans compter pour organiser la mobilisation contre l'épidémie. Chacun de nous se doit de les aider dans cette lutte. Les gestes barrières sont simples : ne soyons donc pas égoïstes ! L'égoïsme, ce serait aussi de jouer avec les peurs, en promettant des mesures inefficaces

part, nous avons choisi de privilégier une coopération européenne et internationale accrue, dans le but d'apporter une réponse collective appropriée. C'est le partage d'informations et d'expériences entre États qui permet de lutter efficacement contre la maladie Cette crise sanitaire appelle également des réponses en matière économique à l'échelon européen. De ce point de vue, Bruno Le Maire a très justement posé la question d'une relocalisation de certaines industries et filières stratégiques en Europe. C'est l'objectif même de l'ambition européenne industrielle et climatique prônée par le Président de la République. Que compte faire le Gouvernement pour accélérer les négociations avec nos partenaires en la matière ?

prenne ses propres responsabilités, sans céder aux ou à une panique totale, même si l'on comprend les inquiétudes dans les secteurs les plus touchés- nos collègues des départements concernés en ont fait part.

alors que c'était l'inverse voilà quelques semaines -participe à cette dégradation. À l'issue de cette crise, que j'espère prochaine- mais, comme l'a dit Claude Malhuret, Dieu seul le sait ... -, il faudra accompagner la reprise de l'économie, ce qui, certes, aurait été plus facile si les marges de manoeuvre dont disposent nos pouvoirs publics étaient plus élevées.

nécessaires aux patients les plus fragiles. La direction générale de la santé a confié à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de

Les liaisons aériennes et maritimes sont les premiers vecteurs de propagation du virus à l'échelle mondiale. À l'intérieur de nos terres, les lignes ferroviaires, les métros et les RER sont également des zones à haut risque. Nous savons que la propagation du virus se fait à 80 % par contact manuel ou par l'intermédiaire d'un objet contaminé. Aussi les salariés des entreprises de transport et les usagers des transports sont-ils exposés à un risque de contamination particulièrement important. actuellement, les entreprises de transport ne disposent pas de protocoles communs par mode de transport pour limiter le risque. Dans ces conditions, nous savons que de nombreux salariés feront le choix d'exercer leur droit de retrait, si l'approvisionnement en masques de protection FFP2 et en gels hydroalcooliques n'est pas assuré dans la durée. Au-delà de l'aspect sanitaire, les conséquences économiques pour certaines compagnies terrestres, maritimes ou aériennes se mesurent déjà en centaines de millions d'euros. Monsieur le ministre, nous ne pouvons faire l'impasse sur la prévention du risque d'infection dans les transports, car cela conduirait à la paralysie de notre pays. Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il pour garantir une protection efficace aux salariés des entreprises de transport en commun ?

Ce soir, avec 3 000 personnes infectées et plus de 100 morts, nos voisins italiens viennent de décider la fermeture des écoles et des universités jusqu'au 15 mars dans tout le pays. Sans parler des mesures prises par Israël. En France, nous considérons manifestement ces mesures comme excessives. Alors, expliquons pourquoi. Tel est, je crois, l'intérêt d'un tel débat. Dans mon département, dix nouveaux cas ont été diagnostiqués aujourd'hui. J'ai le

Seule une communication régulière du Gouvernement à votre niveau et de votre part me paraît pouvoir répondre aux inquiétudes de nos compatriotes. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, je vous confirme que, derrière chaque décision de politique publique que je prends comme ministre, il y a des blouses blanches : toutes les décisions sont concertées. Personne ne peut se dire lui-même expert. Précédemment, l'une de vos collègues-

par des faits avérés, démontrés et publiés. Nous travaillons en concertation avec l'ensemble de nos collègues dans le monde entier pour prendre des décisions raisonnables. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont simples à comprendre,

Deromedi. Monsieur le président, monsieur le ministre, en dehors de la Chine, 79 pays ont signalé des cas. Les cinq continents sont concernés. Nos compatriotes établis en Chine, à Singapour, en Corée du Sud, en Iran, en Italie et dans bien d'autres pays, subissent les restrictions qui y sont imposées. Certains ont fait le choix d'être rapatriés. D'autres sont restés, par solidarité avec les habitants du pays qui les accueille ... Certains lycées français ferment leurs portes par mesure de précaution. L'activité économique est ralentie et certains de nos compatriotes sont soit licenciés, soit priés de prendre leurs congés sans savoir jusqu'à quand. C'est dans ces périodes que l'on se rend compte de l'importance du rôle de nos conseillers des Français de l'étranger, qui agissent conjointement avec les ambassadeurs et les consuls pour prendre en mains la sécurité sanitaire de nos compatriotes. ailleurs, le classement des pays à risques est surprenant. Certains pays, tels que Singapour, font l'objet d'une stigmatisation, alors qu'ils sont transparents, à l'inverse d'autres qui ne publient pas leurs chiffres et ne font donc pas l'objet de restrictions. Le 28 février, nos compatriotes inscrits sur le dispositif Ariane ont reçu un message relatif au coronavirus indiquant : « À ce stade, plusieurs centaines de décès sont recensés à Singapour, le bilan étant en constante augmentation. »

Certes, un démenti a été effectué, mais le mal était fait. Le climat de psychose ainsi créé aura sans nul doute laissé des conséquences sur nos relations diplomatiques et commerciales. il est indispensable de réactualiser régulièrement la liste des pays à risques et le stade de développement de l'épidémie en tenant compte de l'évolution du nombre de cas toujours actifs. Par exemple, Singapour, qui a été classé « orange » avec 112 cas et qui n'en a plus que 33 aujourd'hui, est toujours classé « orange ». Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures sont envisagées pour soutenir nos compatriotes établis hors de France et obtenir que la liste des pays à risques soit réajustée régulièrement ?

Mon interrogation porte sur les conditions de prise en charge des malades identifiés dans les départements ruraux comparables à l'Aisne, éloignés d'un centre hospitalier universitaire. La situation de notre pays exige unité, coordination, totale transparence et confiance dans notre système de santé. Toutefois, nous savons tous que notre système hospitalier est en difficulté, parfois déstabilisé. Pouvez-vous nous assurer, monsieur le ministre, que dans tous les départements, y compris ceux qui ont les structures hospitalières les moins développées, les moyens humains et matériels sont bien en place pour accueillir les premiers malades et faire face, peut-être prochainement, au stade 3 de l'épidémie Ma seconde question porte, en miroir, sur la médecine de ville, appelée, pour ne pas engorger les hôpitaux, à prendre en charge les malades atteints par des formes bénignes. Les médecins généralistes sont prêts à assumer cette responsabilité. Néanmoins, ceux avec lesquels j'étais en contact ce matin, au-delà des nombreux mails d'information qu'ils ont reçus, n'étaient toujours pas destinataires

Deux arrêtés préfectoraux pris le lundi 2 mars ont restreint fortement les activités et l'ouverture des lieux publics dans le département jusqu'au 14 mars, en lien avec les mesures sanitaires prises par le Gouvernement : interdiction de tout rassemblement public, fermeture des cinémas, des théâtres, des discothèques, des administrations et, sur la zone du, des établissements scolaires, des marchés et des piscines, Tout d'abord, si ces mesures visent à contenir au maximum l'épidémie- on ne peut que s'en réjouir -, nous sommes confrontés à un certain nombre d'incompréhensions légitimes de la part de nos concitoyens. Pourquoi fermer un marché, alors que le centre commercial bondé est ouvert ? Pourquoi les boîtes de nuit sont-elles fermées, mais pas les bars de nuit ? Pourquoi la piscine de Vannes est-elle ouverte, mais pas celle de Lorient ?

appels comptabilisés hier au centre hospitalier de Vannes, soit trois fois plus qu'une journée normale. Cette surcharge a évidemment une incidence sur la prise en charge des vraies situations d'urgence. Nous nous acheminons sans aucun doute

Pour autant, je vous rejoins sur le fait que certaines décisions locales paraissent manquer par endroits de clarté. Ce sujet a été abordé ce matin au cours du Conseil national de défense auquel j'ai participé, en présence du Président de la République et du Premier ministre. Je peux vous informer qu'une instruction sera

Alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens n'a jamais été aussi bas en Chine, le berceau de l'épidémie, les autres pays voient la maladie se propager comme une traînée de poudre. En France, plus de 285 cas sont confirmés et quatre personnes sont décédées. Dès l'annonce, par l'OMS, des premiers cas suspects dans la ville de Wuhan au début du mois janvier, le consortium REACTing a été mobilisé pour assurer le partage d'informations scientifiques et coordonner l'effort de recherche français. Pour rappel, le consortium REACTing est un consortium multidisciplinaire rassemblant des équipes et laboratoires d'excellence, afin de préparer et coordonner la recherche pour faire face aux crises sanitaires liées aux maladies infectieuses émergentes. Pour aller encore plus loin, je vous indique que le consortium a identifié plusieurs axes de recherche : le suivi et la modélisation de l'épidémie, la caractérisation du virus, la mise en place et l'amélioration des techniques de diagnostic, ainsi que les pistes thérapeutiques.

Cette épidémie touche aujourd'hui tous les continents et, partout dans le monde, les scientifiques spécialisés en épidémiologie étudient son évolution et son éventuelle mutation. Monsieur le ministre, vous avez montré votre volonté d'accompagner les chercheurs français. Pour autant, sachant que cette épidémie ne connaît pas de frontière, pouvez-vous attester d'une volonté commune, à ce jour, de développer une coopération médicale européenne, voire mondiale, pour pallier la propagation de cette épidémie ? La parole

Le séquençage du génome du coronavirus a été réalisé en France par l'Institut Pasteur, qui travaille, avec d'autres acteurs de la recherche, au développement d'un vaccin. On le sait, ce vaccin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la protection des médecins généralistes, qui déplorent le manque de considération des autorités de santé. Or nous allons entrer dans une phase où l'essentiel de la prise en charge va reposer sur eux, avec un report de l'hôpital vers la médecine de ville. Celle-ci sera en première ligne pour gérer l'épidémie. Les consignes restent peu claires sur la façon de prendre en charge les malades sans risquer d'être contaminé ou de propager ensuite le virus.

En outre, les médecins libéraux ne savent pas précisément à combien de masques ils ont droit, et la distribution a tout juste commencé hier. Ils veulent être protégés avec certitude, mais, à ce jour, on ne peut exclure les contaminations de médecins sur le terrain. rien ne garantit l'entière efficacité des « masques bavettes » pour protéger du coronavirus. Ce choix repose sur l'avis de sociétés savantes et sur un article du (JAMA) dont l'étude, certes intéressante, a concerné un nombre très insuffisant de cas pour mettre en évidence une preuve scientifique irréfutable. De plus, l'étude portait sur le virus de la grippe, dont la létalité reste très inférieure à celle qui est liée au coronavirus. Les médecins doivent donc avoir l'assurance que ce changement de doctrine n'est pas adossé à une réalité pratique, celle de la pénurie de masques FFP2, d'autant plus que, lors de l'épisode de la grippe H1N1, je le rappelle, ces masques-là qui leur avaient été distribués. Ils ont besoin d'un discours de vérité et de transparence concernant cette pénurie. C'est une question de confiance entre eux et les pouvoirs publics. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où en sont les décisions prises avec les industriels français ? Des masques FFP2 sont-ils prévus pour eux, une fois la pénurie hospitalière compensée ? Et dans combien de temps ?

j'ai reçu les conclusions avant-hier -par la Société française d'hygiène hospitalière ainsi que par la Société française de santé publique, cette solution des deux barrières

Magras. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à ce jour, Saint-Barthélemy n'enregistre qu'un seul cas confirmé d'infection au coronavirus. Pour autant, sur notre île, où chacun ou presque se connaît, l'anxiété peut vite grandir. Par ailleurs, le tourisme constituant l'activité dominante de l'économie, l'île est particulièrement exposée, du fait d'une fréquentation touristique cosmopolite et de sa médiatisation à une échelle internationale. Saint-Barthélemy, comme vous le savez, est en situation de double insularité, dès lors qu'elle est reliée à Saint-Martin et à la Guadeloupe en matière sanitaire. La chaîne de prise en charge doit donc être pensée pour s'adapter à ce contexte particulier. Dans cette situation de risque, la réduction au maximum des délais d'acheminement des prélèvements de dépistage et des délais d'évacuation sanitaire, en cas de nécessité de prise en charge hospitalière, sont les deux leviers majeurs pour permettre de prévenir la diffusion du virus et rassurer la population. Ainsi, les résultats d'analyses biologiques doivent pouvoir être obtenus dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Monsieur le ministre, des moyens ont-ils été déployés pour garantir ce délai ? De même, les moyens sont-ils mis en oeuvre pour qu'il soit possible, si l'évolution de la situation le requérait, de gérer plusieurs évacuations sanitaires simultanées ou très rapprochées vers les centres hospitaliers de la région ?

dans toute la Chine, en Asie ensuite, et désormais dans de nombreux pays où le virus s'est propagé. Dans tous ces pays, les Français de l'étranger ont pu compter sur le précieux soutien du ministère des affaires étrangères, qui a su répondre efficacement aux nombreux défis posés par la propagation de l'épidémie. Je pense particulièrement à l'évacuation de nos compatriotes présents à Wuhan et tiens ici à remercier le personnel de nos ambassades et de nos consulats de leur engagement. Cependant, l'inquiétude parmi la communauté française est multiple et forte. Elle porte notamment sur la scolarisation des enfants, car à ce stade, de nombreux établissements français à l'étranger sont fermés à la demande des autorités locales.

Dans ce contexte, la question du bon déroulé des examens soulève déjà de nombreuses inquiétudes. Les personnels français s'interrogent également sur les mesures qui seront prises en cas d'aggravation de la situation sanitaire- peut-être un rapatriement La stabilité financière des établissements scolaires est aussi une source de préoccupation, car il est fort possible que de nombreuses familles ne puissent plus contribuer financièrement au fonctionnement de ces établissements.

Depuis le début de la crise, l'AEFE a instauré, avec le soutien du CNED et la mobilisation de toutes les équipes enseignantes locales, un dispositif d'enseignement à distance, grâce auquel les élèves de toutes sections ont pu travailler au moins trois heures par jour jour et une déscolarisation massive a pu se poursuivre jusqu'à présent, avec des mesures d'accueil en présentiel lorsque c'était possible. Une extension durable de la crise du coronavirus à d'autres pays aura des conséquences économiques potentiellement lourdes pour les établissements d'enseignement. Il faudra donc y porter une attention particulière, que le fonctionnement du réseau est déjà très perturbé en Asie. Le Quai d'Orsay est en relation permanente avec le ministère de l'éducation nationale pour régler tous les différents problèmes rencontrés.

dans de nombreux secteurs économiques. Le premier domaine immédiatement touché est celui du tourisme, avec des conséquences sur les hôtels-restaurants, les entreprises d'événementiel, les traiteurs, particulièrement dans les grandes villes, où les événements d'ampleur ont été interdits. Au-delà de l'annulation de ces événements, une véritable psychose s'est installée et les annulations de séminaires, petits salons, événements d'entreprise dépassent très largement le seul cadre des décisions gouvernementales ou préfectorales. Sur ce secteur du tourisme, l'Europe a déjà perdu 2 milliards d'euros depuis le début du mois de janvier, selon la Commission européenne. Mais, en France, c'est un secteur particulièrement fragilisé, ayant subi depuis plusieurs années des chocs à répétition : d'abord les retombées des attentats,

avec des reports de charges ou du cautionnement de besoins de trésorerie. Mais, au-delà de ces mesures utiles, il faudra cette fois plus et, surtout, tout de suite. Il faut suivre chacune des entreprises individuellement, car il est à craindre qu'elles ne disposent plus maintenant de la résilience nécessaire pour absorber ce nouveau choc, le troisième en deux ans. Ainsi, c'est à un véritable effondrement immédiat auquel nous assistons.

depuis le 3 mars au ministère de l'économie. Elle permet d'obtenir toutes les informations nécessaires sur la situation économique du pays en temps réel. Le but est de mieux gérer l'impact de la crise sanitaire sur notre économie, en prenant, au quotidien, les décisions qui s'avèrent nécessaires. En outre, nous allons reporter

Il est reconnu et documenté que l'hébergement en institution peut favoriser la diffusion des virus. Le Covid-19 ne fait et ne fera pas exception. Les personnes âgées figurent parmi celles qui sont les plus exposées à un risque, de par leur vulnérabilité aux infections respiratoires aiguës, mais aussi le profil de comorbidité présenté par certains sujets. Je rappelle que le virus de la grippe reste le premier facteur de mortalité dans les établissements.

des autres établissements, dans ses dernières recommandations adressées aux professionnels du secteur médico-social, votre ministère les incite à identifier les salariés revenant des zones à risque. Dans ces cas de figure, le personnel est invité à ne venir travailler qu'après la période de quatorzaine ou à voir ses activités réorganisées pour ne voir ses activités réorganisées pour ne pas être mis en contact avec des personnes vulnérables. Ainsi, dans un contexte général d'activité déjà particulièrement tendue, on ne peut pas ne pas penser aux résidents. âgées (Synerpa) envoyait aux établissements un rappel des mesures générales à appliquer concernant la continuité d'activité.

mon intervention, à saluer le travail remarquable de l'ARS et de son directeur général, qui a été en liaison permanente avec les élus, mais aussi du personnel hospitalier, des services de l'État et des collectivités concernées. C'est tous ensemble que nous parviendrons à apaiser les esprits, à informer au mieux pour avoir les gestes et attitudes appropriés à chaque stade de la propagation de ce virus.

l'un des parents doit se mettre en arrêt maladie pour garder son enfant. Cet arrêt est normalement géré par les médecins de l'ARS. Or ces derniers, sur-sollicités, sont difficilement joignables. Certaines personnes se tournent alors vers le SAMU, ce qui n'est pas gérable sur le long terme. Il serait donc souhaitable que les médecins libéraux puissent délivrer ces arrêts de travail, au moins de manière temporaire, pour décharger l'ARS et le SAMU. De ce fait, il faut alerter sur le risque de saturation du 15. Le SAMU, dans certaines zones, pourrait être complètement débordé, et n'oublions pas que les autres malades ont toujours besoin de soins d'urgence, en cas d'infarctus par exemple Il serait également profitable pour les ARS de créer des numéros verts zonaux, c'est-à-dire par zone de défense, la Haute-Savoie se trouvant à ce titre dans la zone Sud-Est. Cela permettrait à des médecins libéraux volontaires de répondre aux questions et de réexpliquer les bonnes pratiques à observer pour éviter la propagation du virus. Les ARS seraient alors partiellement déchargées.

Monsieur le ministre, si l'épidémie engendre son lot d'incertitudes et de questionnements, il est en revanche une certitude, c'est que, à l'instar du corps médical, des personnels hospitaliers, les élus et, singulièrement, les maires se trouvent en première ligne. Dans les communes touchées, ou qui le seront demain, les maires, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, sont amenés à faire respecter les interdictions préfectorales de rassemblement et les fermetures des lieux recevant du public, à commencer par les par les écoles, les marchés, jusqu'aux équipements sportifs. Je pense aussi à la question particulière des Ehpad, lieux de vie et d'échanges avec l'extérieur, dont les résidents constituent la partie de la population la plus exposée aux risques du coronavirus. Le niveau 2 d'alerte ayant été déclenché, nous devons tous anticiper la mise en place du troisième palier. Celui-ci sera sans doute assorti de mesures plus drastiques, qui auront des conséquences sur le quotidien de nos concitoyens. Ces conséquences nourriront un inévitable sentiment de frustration si le bien-fondé mal accepté et si aucun interlocuteur de proximité n'est capable de les justifier avec tact et pédagogie. Dans une crise comme celle à laquelle nous nous préparons, la crédibilité de la parole publique et le respect des des décisions prises par les autorités sont primordiaux. Au contraire, la défiance risquerait de désarmer la lutte contre l'épidémie. Heureusement, ces interlocuteurs de terrain existent : ce sont les 35 000 maires

municipal et certains conseillers municipaux de la commune voisine, car il m'a semblé tout à fait naturel, dans le cadre de mon premier déplacement sur le terrain en zone d'activité virale, d'aller à la rencontre des élus locaux. Ce sont eux que la population interpellera,

Elle nécessite une grande réactivité, ce qui n'est pas toujours facile. À titre d'exemple, monsieur le ministre, conformément aux recommandations de votre ministère, nos concitoyens modifient leurs comportements en vue de contenir la propagation du virus. Conséquence fâcheuse, les solutions hydroalcooliques viennent désormais à manquer en de nombreux points du territoire. mondiale de la santé (OMS) a publié en ligne un guide pour aider les particuliers à élaborer leur propre gel désinfectant, ce qui pose question sur la conformité, l'innocuité, la revente, etc. monsieur le ministre, que nos pharmaciens ont les capacités matérielles de préparer de telles solutions en officine, et ce très rapidement. Vous savez également qu'ils ne peuvent le faire en raison de contraintes légales. En effet, ces solutions hydroalcooliques ne font pas partie des préparations officinales au sens de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. À son article L. 3131-1, ce même code vous offre pourtant la possibilité de prendre des mesures d'urgence en cas de menace d'épidémie. Dérogatoires, elles pourraient autoriser les pharmaciens à commercialiser leurs propres préparations sans délai. Au-delà de la question des solutions hydroalcooliques, je me dois aussi d'attirer votre attention sur la réquisition des masques anti-projections. Premiers relais de cette distribution nationale ciblée à destination des professionnels de santé, les pharmaciens ne peuvent pas en bénéficier eux-mêmes. Au contact permanent de leur clientèle, ne sont-ils pas, pourtant, exposés au même titre que les autres professionnels de santé ? Qu'en serait-il de cette distribution si ceux qui sont chargés de l'organiser étaient atteints, faute de protection ? Monsieur le ministre, envisagez-vous d'accorder aux pharmaciens, dont le réseau maille le territoire, les moyens matériels et réglementaires appropriés dans cette lutte contre le virus ? La parole

et les patients n'ont qu'à pousser leur porte pour avoir un accès direct à un professionnel de santé. Je pense qu'il faut utiliser à plein ce réseau dans le cadre particulier de cette épidémie. Les pharmaciens peuvent fabriquer ces gels hydroalcooliques, ce qui éviterait la pénurie que nous connaissons aujourd'hui. Par ailleurs, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question, portant sur le fait que les pharmaciens n'ont pas accès aux masques de protection, alors même qu'ils sont censés les distribuer aux professionnels de santé et qu'ils sont eux-mêmes en première ligne face aux malades. Mes chers

La séance est levée.